Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 26 janvier 2017, le texte d'une décision statuant sur la conformité à la Constitution de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Cette loi, que je considère comme très importante, régit les rapports entre les communes, l'État et un certain nombre d'organismes pour l'entretien des ouvrages d'art situés au-dessus ou en dessous de routes communales : cela concerne les autoroutes, les canaux, les voies ferrées. Pour ce qui est des ouvrages d'art anciens, la loi avait prévu qu'un recensement soit effectué afin qu'une solution définitive soit proposée au plus tard en 2018.

n'a pourtant pas répondu aux besoins pressants de l'institution judiciaire, qui traverse une crise grave. Ce constat, vous avez bien voulu le partager avec nous lors de votre nomination aux fonctions de ministre de la justice et de garde des sceaux.

Les conséquences sont à ce jour considérables, car les choix de ce gouvernement ont été portés par un dogmatisme à toute épreuve, fondé le seul objectif de désencombrer les prisons,

Notre justice est marquée depuis plusieurs décennies par une augmentation des contentieux, tant en matière civile et pénale qu'en matière administrative, et par un encombrement avéré. Nous le savons, les magistrats assument leur rôle, et nous leur redisons toute notre confiance, mais notre justice n'a plus aujourd'hui les moyens d'accomplir sa mission et, surtout, d'être crédible et respectée par les justiciables. Ce que les Français ne supportent plus, ce sont bien sûr les lenteurs liées à l'engorgement des tribunaux, mais surtout la non-exécution des peines prononcées en matière pénale. Il est urgent de mettre fin à cette situation, situation, car nous ne pouvons accepter cette remise en cause. Vous avez voulu porter l'ambition d'une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice pour nos concitoyens. Pourtant, la défiance des Français envers la justice est actuellement grande : 64 % de nos concitoyens La seule certitude aujourd'hui, c'est que notre système judiciaire ne passera pas le XXIsiècle si les décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant sont maintenues et si nous ne modifions pas fondamentalement les choses. Rien n'est pourtant plus éloigné de la réalité que les projets qui ont été soutenus jusqu'à présent. Le meilleur exemple, le plus symbolique, est celui de la contrainte pénale. Ce que je me permets de qualifier de « Canada Dry de l'alternative à la prison » est né dans la confusion pour survivre dans le trouble. Les magistrats ne la prononcent pas parce qu'ils doutent eux-mêmes de son efficacité. Alors oui, pour des raisons très pragmatiques, et non pas idéologiques, comme nous l'avons entendu dire lors de la réunion de notre commission, nous souhaitons la supprimer. Notre objectif rejoint celui des professionnels : rendre à la justice son efficacité. C'est bien tout le sens de la proposition de loi que mes collègues cosignataires

doit être efficace pour redonner du sens à la peine, ce qui impose notamment de lui redonner des moyens à hauteur de ses besoins. Rendre son efficacité à la justice permettra de rendre une justice plus protectrice de nos concitoyens afin que soient assurées, en tout lieu du territoire, la sûreté des biens et des personnes, mais aussi la protection des droits et des libertés. Nous proposons donc de systématiser et d'accélérer la mise en oeuvre de la sanction afin de redonner leur valeur d'exemplarité aux décisions de justice et du sens à la peine. La loi pénale doit avoir une vocation sociale dissuasive. C'est pourquoi nous proposons de réinstaurer les peines planchers. Ne criez pas au loup trop rapidement, chers collègues : nous les avons modernisées et adaptées au XXIsiècle ! Elles ne pourront concerner que les crimes et délits passibles de plus de cinq ans d'emprisonnement. Les peines minimales sont un dispositif garantissant une plus grande sévérité à l'égard des récidivistes. Si ces peines ne permettaient pas l'individualisation des peines, comme nous l'avons trop souvent entendu dire, le Conseil constitutionnel l'aurait censuré dès 2007 La protection des droits, à laquelle le Sénat est constamment attaché, est fondamentale dans un contexte où le pouvoir régalien de l'État déploie toute sa mesure, mais elle doit être fondée sur des rapports de réciprocité. Or ces rapports sont aujourd'hui asymétriques. C'est pourquoi il est nécessaire de nous interroger sur la part de chacun dans l'exécution de la peine et la prévention de la récidive. L'automaticité des réductions de peines, à échéance fixe, rompt l'effectivité des décisions de justice. Cette rupture est tragique pour les victimes, on le comprend aisément, mais elle est fatale aussi pour les délinquants. Les taux de récidive, que le ministère de la justice a grand mal à nous communiquer, sont sans équivoque. Comment un délinquant, entré souvent très jeune dans la spirale infernale, peut-il comprendre que son acte est grave si la peine qu'il purge est réalisée selon des modalités définies par le temps ? Or le fondement actuel des réductions de peines est bien celui du temps, un droit octroyé par provision. Nous vous proposons d'inverser cette logique, de revisiter l'accès au bénéfice de la réduction de peine, en posant le principe qu'elle est non pas un droit acquis, mais une faveur octroyée en considération des gages donnés par le condamné de sa volonté de réinsertion. Nous sommes convaincus que c'est notamment par ce nouveau contrat social que nous inverserons la spirale de la récidive. Ce changement de paradigme sera accompagné de la mise en place d'un tribunal de l'application des peines qui, collégialement, adaptera les décisions en fonction des risques potentiels liés à la libération anticipée d'un individu et qui permettra d'avoir un regard différencié sur la personnalité du délinquant mis en cause.

C'est pourquoi, sans remettre en cause la nécessité d'étendre le parc pénitentiaire, il nous est apparu intéressant de proposer la création de centres de rétention pénitentiaire à sécurité adaptée, à raison de la peine ou du profil de la personne concernée, dans l'unique objectif de lutter contre la récidive. Mes chers collègues, nous ne vous présentons pas une législation de plus alors que les professionnels et les justiciables étouffent sous l'accumulation grandissante des normes.

pénale. Cette proposition de loi trouve sa source dans une constatation qu'il serait irresponsable de négliger : la crédibilité de la justice pénale ne cesse de s'éroder dans l'opinion publique. Or on ne peut pas prétendre revaloriser la justice sans se préoccuper de la valorisation de son image. On ne peut pas vouloir conforter l'autorité judiciaire sans préserver l'adhésion à ses décisions. on ne doit pas lui enjoindre de n'être que l'expression de la au premier motif que son indépendance est protectrice de l'État de droit. La justice, dont l'indépendance doit être garantie, est, proclame-t-on, rendue au nom du peuple français. Nos concitoyens exigent légitimement d'être écoutés. Cependant, ils ne sont pas sourds à l'énonciation des faits, pourvu que ceux-ci soient vérifiés, et ils ne répugnent pas à adhérer aux règles fondamentales de notre droit, pourvu qu'elles soient justifiées et expliquées. Or, précisément, sans bouleverser ou affaiblir les grands principes de notre droit pénal, il est possible de satisfaire les attentes de nos concitoyens en préservant l'autorité judiciaire de toute atteinte

ont à juste titre et opportunément suscité une réflexion sur plusieurs progrès législatifs tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale. L'ensemble des auditions, plus constructives que critiques, les contributions citoyennes recueillies sur l'espace participatif que j'ai ouvert sur ces questions l'attestent également.

Cette affirmation, en trouvant un écho réel dans nos travaux au travers de modifications législatives précises, permettra de répondre aux incompréhensions de celles et ceux qui, admettons-le, n'acceptent pas ce qu'ils ressentent, sur un plan général, comme l'expression affaiblie de la justice et, dans leur vie quotidienne, comme une négation de leur droit à la sécurité. À travers plusieurs dispositions pour renforcer la certitude de la peine, la proposition de loi tend à améliorer la procédure pénale tant dans sa phase présentencielle que dans la phase de jugement. Cette proposition de loi vise ainsi, pour faciliter la répression des infractions, à mieux encadrer la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites, à renforcer les prérogatives du parquet dans la conduite des enquêtes et pour les placements en détention provisoire, à consacrer de nouvelles garanties dans la phase de jugement. Elle conforte aussi la réponse pénale et son exécution par la menace d'une sévérité renforcée, par la certitude de l'effectivité de la sanction au travers d'un meilleur encadrement du régime d'application et d'exécution des peines. la proposition de loi contient des mesures aménageant la législation contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et renforçant la protection des mineurs victimes d'infractions. La commission des lois a approuvé les orientations du texte, estimant que nombre de ses dispositions étaient utiles. Elle s'est donc attachée à l'examen de leur constitutionnalité, de leur conventionnalité et de leur cohérente et efficace intégration dans notre État de droit. Elle a ainsi été conduite à retenir des améliorations, certaines purement rédactionnelles, pour qu'il ne soit pas, même indirectement, porté atteinte au champ d'application du principe d'opportunité des poursuites ou à l'effectivité du principe d'individualisation des peines. peines. Je tiens surtout à attirer votre attention sur le résultat fondamental des orientations et de la voie choisies pour assurer un solide équilibre : la commission des lois a retenu le constat sociologique des auteurs de la proposition et l'objectif des mesures qu'elle contient en préservant l'absolu pouvoir du juge. le juge devra plus encore que précédemment motiver ses décisions, mais c'est précisément ainsi qu'il légitime et renforce la justice qu'il rend au nom du peuple. Nous ne pouvons pas négliger ce que nous entendons sans cesse dans tous les territoires, dans toutes les couches de la société quels que soient les âges, dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Prenons l'instauration des peines planchers. Tous les propos excessifs peuvent, je vous l'assure, être écartés. Notre concitoyen peut demander que celui qui a été condamné plusieurs fois, qui a bénéficié de mesures alternatives aux poursuites, de sursis successifs, d'accompagnements, de libérations anticipées, qui a été averti, voie sa prochaine peine affectée d'un minimum. Il est même parfaitement légitime à le souhaiter quand, s'adressant à nous, il admet : « Législateurs, vous m'avez enseigné le principe de la nécessaire individualisation des peines et maintenant j'y adhère ; je comprends pourquoi la peine plancher que je réclamais ne peut en aucun cas être automatique ; je conçois, monsieur le juge, que vous ayez écarté son application, mais dites-moi pourquoi

Les faits, c'est montrer que les magistrats ne sont pas laxistes. Le taux de réponse pénale est actuellement supérieur à 90 %. Les peines prononcées sont en moyenne plus lourdes. Alors que le nombre d'affaires susceptibles de poursuites est en diminution, on constate une aggravation des peines prononcées qui se traduit par un recours plus important, tant en proportion qu'en valeur absolue, à la peine d'emprisonnement. Entre 2011 et 2015, le nombre de peines d'emprisonnement ferme a augmenté de 10 %. Au mois de juillet 2016, plus de 69 000 personnes étaient détenues, soit le maximum jamais atteint. Au cours de cette même année, la population carcérale a progressé de 3,3 %, soit plus que l'augmentation de la population française ou la hausse de la délinquance. Les faits, Les faits, c'est aussi prendre en compte les propos de la grande majorité des magistrats entendus qui disent ne pas appliquer la contrainte pénale parce qu'ils peuvent utiliser la mesure proche et plus éprouvée du sursis avec mise à l'épreuve. La pédagogie, c'est expliquer que toute remise en liberté sans condition, ni surveillance ou accompagnement ne participe pas à la réinsertion mais augmente le risque de récidive. La pédagogie, c'est convaincre que, dans le traitement de la délinquance, la répression est nécessaire, mais pas toujours suffisante. Enfin, revenant aux réflexions directement inspirées par la proposition de loi de François-Noël Buffet, de Bruno Retailleau et des autres cosignataires, mérite de nous inviter, sans les clore, à deux débats futurs incontournables pour répondre aux incompréhensions et aux attentes de nos concitoyens : d'une part, la suppression définitive de toutes les mesures de remises automatiques de peine au profit d'un régime unique

organiser un autre épilogue aux audiences à l'issue desquelles l'auteur condamné à une peine privative de liberté quitte libre l'enceinte judiciaire aux côtés de la victime. Un journal du soir, et plus précisément d'hier soir, fournit quelques exemples. On pourrait en citer de bien plus humainement inacceptables. Quelles que soient nos convictions sur ces sujets complexes, il est sociologiquement irresponsable de les traiter avec complaisance ou condescendance Mais, pourquoi le nier ? tout ce qu'il reste à faire, toutes les mesures que nous prendrons auront pour effet, nonobstant le pouvoir d'appréciation réservé et ultime des juges, de nécessiter des investissements importants en matière d'établissements pénitentiaires et l'octroi de moyens supplémentaires. il ne s'agit pas d'une nécessité récente attribuable à cette proposition. Rappelons-nous le plan mis en place en ce domaine par notre collègue Michel Mercier lorsqu'il était ministre de la justice, qui fut quasiment immédiatement abandonné par son successeur.

les sénateurs, dans, Jean-Paul Sartre fait dire à l'un de ses protagonistes que « tous les moyens sont bons, quand ils sont efficaces ». La notion d'efficacité constitue le coeur du texte qui nous réunit aujourd'hui. La définition

simplicité ? Est-ce la cohérence ? Cet exercice de définition n'a rien d'oiseux, bien au contraire. Lorsque l'on choisit des mots, il faut le faire en connaissance de cause, et c'est tout l'enjeu de notre débat. La proposition de loi qui est soumise à notre discussion contient plusieurs mesures, dont l'objectif explicite serait d'améliorer l'efficacité de notre justice pénale. Le texte prévoit ainsi de rétablir des peines minimales pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans ; de restreindre le quantum des peines aménageables ; de renforcer les règles de révocation des sursis ; de restreindre le champ d'application de la confusion de peines ; de supprimer la contrainte pénale et la libération sous contrainte. Toutes ces mesures, quand on les analyse les unes après les autres, ont pour point commun de chercher à durcir la répression. Est-ce efficace ? Je ne le crois pas. Par exemple, une part notable des dispositions initiales de la proposition de loi avaient surtout pour conséquence essentielle de rigidifier, voire d'alourdir le fonctionnement de la justice pénale. Je me félicite donc du fait que la commission des lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, ait supprimé purement et simplement quatre articles du texte initial. Je relève aussi avec intérêt qu'elle a décidé d'en réécrire plusieurs autres, intégralement.

mesure soulevait évidemment une difficulté d'ordre constitutionnel liée à l'absence de révision du statut du parquet, une révision qui, soit dit en passant, a été proposée par le Gouvernement, mais que le Sénat

ni efficace au sens de « plus rapide », ni efficace au sens de « plus simple », ni efficace au sens de « plus cohérent ». Non seulement ce texte n'apporterait pas d'efficacité mais, de surcroît, j'en suis convaincu, il nuirait à l'efficacité de la justice pénale. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut soutenir cette proposition de loi. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas la conception que nous nous faisons de l'efficacité. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de la justice pénale. Revenons à l'étymologie du terme « efficacité ». Émile Littré nous renseigne à merveille : l'efficacité vient du latin, qui signifie « force », « vertu ». Donner plus de force à la justice pénale ? Mais nous l'avons fait ! Nous ne cessons de le faire depuis 2012 ! De ce point de vue, nous sommes unanimes : l'efficacité de la justice, qu'elle soit pénale ou civile, réside avant tout dans ses moyens.

Je l'ai dit et je ne cesse de le répéter : le ministère de la justice souffre d'une vraie difficulté, à savoir son budget. Vous le connaissez, vous l'avez discuté et vous avez noté que des avancées objectives ont été obtenues. En 2016, le dégel anticipé de 107 millions d'euros au profit des juridictions a permis d'éviter des ruptures de paiement. En 2017, l'ouverture de 40 millions d'euros par décret d'avance va permettre d'augmenter massivement les dépenses consacrées aux juridictions. Tout cela a un effet directement mesurable. Vous avez probablement participé aux audiences de rentrée dans les TGI et dans les cours d'appel, et vous avez entendu ce qui a été modifié dans l'année. Je citerai simplement deux cas précis. Les arriérés de paiement de la cour d'appel de Rennes étaient de 5 millions d'euros début 2016 ; ils sont aujourd'hui de 800 000 euros. À la cour d'appel de Colmar, ceux-ci étaient de 2,9 millions d'euros au début de l'année 2016 ; ils sont désormais de 430 000 euros. Sur l'ensemble du territoire, le délai de paiement des frais de justice est passé, en un an, de quatre mois à un mois. C'est cela, mesdames, messieurs les sénateurs, l'efficacité de la justice ! Pour 2017, l'effort sera soutenu, avec un budget de 7 milliards d'euros, en augmentation de 4,2 %. Cela aussi contribuera à l'amélioration de l'efficacité. Après avoir redressé la situation des frais de justice, j'entends m'atteler aux dépenses de fonctionnement et d'investissement. À cette fin, le budget de 2017 augmente de 10 % les crédits de fonctionnement des services judiciaires et de 28 % les crédits immobiliers. Enfin, pour que ces majorations de crédits puissent rapidement être perçues par les juridictions, le Premier ministre a accepté de lever totalement le gel concernant ces dépenses. Cela correspond à un montant de 40,5 millions d'euros, soit 28,5 millions d'euros de fonctionnement et 12 millions d'euros d'immobilier. S'agissant des recrutements, j'ai déjà eu l'occasion de le dire au Sénat, mais je veux le répéter,

Corrélativement à l'augmentation des moyens, il faut recentrer les magistrats et les enquêteurs sur leur coeur de métier. Il faut aussi améliorer la gestion des contentieux de masse pour lesquels leur intervention apporte parfois une faible plus-value. Il faut encore simplifier la procédure, qui est parfois devenue inutilement formaliste, tout en renforçant les garanties accordées aux justiciables. Tout cela, nous avons commencé à le faire dans la loi de modernisation de la justice du XXIsiècle, dite « J21 », par exemple avec la forfaitisation de certains délits routiers, dont la constatation ne donnait lieu qu'à très peu de contestation et dont la sanction répondait très largement à des barèmes préétablis. Cela encore améliorera l'efficacité de la justice. C'est également ce que nous avons fait avec le plan de simplification de la procédure pénale, qui s'est traduit par des modifications législatives dans la loi du 3 juin 2016, dans des adaptations réglementaires dans le décret de simplification du 7 septembre 2016, et par deux circulaires de simplification des 23 décembre 2015 et 8 septembre 2016. Ces mesures de simplifications concernent ainsi la la possibilité de transmettre des procès-verbaux sous forme électronique ; la simplification de l'exploitation des supports informatiques saisis au cours de l'enquête, dont la copie peut désormais être faite sans la présence d'un OPJ l'extension des possibilités de comparution forcée, en cas de risque de modification des preuves ou des indices, de pressions sur les témoins ou les victimes et de concertation entre les coauteurs ou les complices de l'infraction. Nous avons simplifié l'extension du recours à la visioconférence pour la présentation au juge, afin d'éviter les contraintes liées au transport de la personne interpellée. Nous avons simplifié encore par la création de plateformes de soutien logistique de gestion de la garde à vue, permettant de rationaliser la mise en oeuvre des droits de la personne placée en garde à vue- recherche d'un médecin, contact avec l'avocat choisi, recherche d'un interprète. Nous avons simplifié en modifiant le principe « un acte-un PV », en permettant aux enquêteurs de regrouper plusieurs actes de procédure en un seul procès-verbal. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui a déjà été fait et qui contribuera nécessairement à améliorer l'efficacité de la justice. Nous avons apporté une certaine souplesse dans les procédures, tout en préservant les garanties fondamentales des uns et des autres. Si l'efficacité signifie étymologiquement « force

d'avoir écrit en introduction de votre rapport : « Statistiquement, la justice pénale n'a jamais été aussi répressive. « Le taux de réponse pénale est actuellement supérieur à 90 %. de juillet 2016, plus de 69 000 personnes étaient détenues, soit le maximum jamais atteint. Au cours de la même année, la population carcérale a augmenté de 3,3 %, soit plus rapidement que la population française. « Pourtant, la crédibilité de la justice pénale ne cesse de s'éroder dans l'opinion publique. Si de nombreuses peines sont prononcées, leur exécution, qui répond à un régime devenu particulièrement complexe au gré des réformes, est loin d'être toujours immédiate et effective »- nous y avons travaillé dans le cadre de la mission

faculté. C'est précisément parce que nous croyons que cette mission peut aboutir que nous voulions vous proposer de renoncer à l'examen de ce texte.

j'essaie de vous accompagner ? J'en doute ! Quoi qu'il en soit, puisque vous tenez absolument à ce que cette proposition de loi soit discutée, je ne soumettrai pas ma question préalable à vos suffrages, respectant la tradition républicaine de cette assemblée,

pour que nous abordions aujourd'hui la question des moyens affectés à la justice pour qu'elle soit plus efficace. Ce sera finalement un rapport complémentaire pour notre mission. La

à empêcher le débat sur cette proposition de loi. Je veux aussi remercier M. Jacques Bigot de l'intérêt qu'il porte, par sa participation très active, aux travaux de la mission d'information que nous avons mise en place sur le redressement de la justice, qui en a, il est vrai, bien besoin.

La première consiste à supprimer la contrainte pénale. La contrainte pénale a été introduite dans notre droit sans aucune étude d'impact et elle s'est heurtée non seulement à des questions de principe sur lesquelles nous reviendrons, mais à l'absence totale de moyens pour sa mise en oeuvre. Il était pourtant indispensable, si on raisonne en termes de bon fonctionnement de la justice, d'assortir toute mesure nouvelle en matière pénale de moyens. En supprimant la contrainte pénale, nous libérerons les magistrats et les services d'insertion et de probation d'une charge potentielle qui n'avait jamais été évaluée. La deuxième mesure, c'est le rétablissement des peines planchers,

de ce texte, c'est la suppression des remises de peines automatiques et de l'examen automatique, à un moment de l'application de la peine, de la situation du condamné. Cette charge pour les magistrats de l'application des peines sera donc supprimée. Aussi, vous le voyez bien, loin de porter préjudice à la réflexion sur le redressement de la justice, ce texte, s'il est examiné non pas du point de vue de l'efficacité de la répression pénale, mais du point de vue des moyens de la justice, allège

selon les auteurs de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale que nous examinons aujourd'hui, « la crédibilité de la justice pénale est fortement érodée dans l'esprit de nos concitoyens. Sa lenteur et son laxisme sont décriés. » Face à ce constat sans appel et puisque, je cite à nouveau, l'heure n'est plus à débattre du bien-fondé de ces critiques récurrentes, il y a urgence à offrir des gages d'du fonctionnement de notre appareil répressif, à chacun des maillons de la chaîne pénale. chaîne pénale. » Concrètement, la grande majorité des dispositions soumises à notre Haute Assemblée dans cette proposition de loi tend à supprimer les dispositions introduites par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. La droite sénatoriale avait combattu ce texte, déposé des centaines d'amendements et crié au laxisme de Christiane Taubira, qui le portait. Vous faites donc preuve de cohérence, mes chers collègues, et peut-être aussi d'anticipation ... Porté notamment par M. Bruno Retailleau, coordinateur de campagne du candidat de la droite, ... Et alors ? ... ce texte donne, je le crois, une idée assez précise de ce que défend le candidat François Fillon en matière de justice pénale. Après plusieurs mois de primaires, de débats internes aux familles politiques, ce texte vient nous rappeler les fondamentaux de la droite en matière de politique pénale tout-répressif, tout-carcéral, défiance envers les magistrats et éternel procès des socialistes accusés de laxisme, voire d'irresponsabilité. Puis-je vous rappeler, mes chers collègues, que la conférence de consensus ayant précédé l'élaboration de la réforme pénale, que vous souhaitez aujourd'hui mettre en pièces, avait montré une chose capitale : l'échec patent de la politique pénale menée pendant dix ans ? En matière de récidive notamment, avec les peines planchers, que vous voulez rétablir aujourd'hui, et qui étaient supposées dissuader les récidivistes potentiels. Il s'est avéré que le taux de récidive avait été multiplié par plus de deux, passant de 6,4 % en 2002 à 14,7 % en 2011. Quant au prétendu laxisme de l'autorité judiciaire, laissez-moi vous donner quelques chiffres : le nombre de peines fermes ou partiellement fermes prononcées par les tribunaux correctionnels a crû de 10 % entre 2004 et 2015. Le quantum ferme moyen a, quant à lui, augmenté d'un mois et demi entre 2012 et 2015- 2015- 8,4 mois aujourd'hui -alors qu'il avait baissé de 1,2 mois entre 2004 et 2012- 8,1 mois contre 6,9 mois. Même si c'est peu surprenant, il est toujours regrettable de constater qu'à mesure que les échéances électorales approchent les outrances et les propos démagogiques se multiplient. C'est le groupe écologiste ne votera pas ce texte inique, mais, puisque l'heure est au retour aux fondamentaux, certaines choses méritent, me semble-t-il, d'être rappelées. La justice de notre pays est en difficulté, en grande souffrance parfois, et ce dont elle pâtit en premier, c'est du manque de moyens chronique. Aucune mention n'est faite dans votre proposition de loi sur les moyens que vous comptez allouer à cette réforme, d'un programme pénitentiaire qui devrait être d'une ampleur inégalée pour remédier à l'état de déliquescence dans lequel il se trouve. Soyons pour une fois honnêtes, mes chers collègues, les lois peuvent être toujours plus répressives, si les magistrats n'ont pas les moyens de les appliquer, votre volonté d'éradiquer la délinquance restera un voeu pieux et s'arrêtera à l'affichage que vous souhaitez en cette période électorale, où il faut plutôt montrer ses muscles que réformer vraiment la justice. La parole

le rapporteur, mes chers collègues, j'ai lu, j'ai entendu que ce texte a été préparé dans la perspective de l'alternance. Si tel est bien le cas, le signe envoyé est inquiétant : plus qu'un travail qui prépare l'avenir, vous nous proposez un retour vers le passé. Le texte initial, avant que notre excellent rapporteur ne l'ait profondément modifié, était, je suis obligé d'employer cette expression, un texte de réaction, un texte, au sens propre, de restauration.

! Or tous les chiffres publiés dans le rapport démontrent le contraire. Notre rapporteur a l'honnêteté de le reconnaître. L'Union syndicale des magistrats l'a également souligné. Jamais, la justice pénale n'aura été aussi répressive. Au 1 juillet 2016, 69 375 personnes étaient incarcérées. C'est un record. Entre le 1 janvier 2006 et le 1 juillet 2016, le nombre total de personnes détenues a augmenté de 19 %. Personnellement, je ne me vante pas de ces chiffres, mais ils constituent la réalité : lorsque la gauche est au pouvoir, l'emprisonnement ne baisse pas ; il augmente, et ce en dépit d'une politique pénale qui a multiplié les peines alternatives. Faut-il alors, par dogme, renouer avec le fil rouge des années Sarkozy ? Répondre systématiquement à l'émotion causée par une nouvelle loi toujours plus répressive que la précédente, toujours plus favorable à l'incarcération, toujours plus aveugle sur les causes de la récidive et le travail de réinsertion du détenu ? Votre programme est un long pensum de redites : des peines planchers, une réduction du quantum des peines aménageables, un abaissement des seuils d'aménagement des peines, le refus de considérer la surveillance électronique comme une peine privative de liberté ... La liste n'est pas exhaustive, j'y reviendrai. Pour permettre Pour permettre cette restauration, il vous fallait bien réidentifier un obstacle, l'obstacle qui vous empêche de transformer un discours à la population en un mandat de dépôt.

en plaçant au-dessus de lui des peines automatiques, en l'enfermant dans un champ d'amendes forfaitaires, en l'obligeant à révoquer le sursis simple ou bien en le contournant par le référé-détention.

Il l'a fait à sa manière, avec beaucoup de finesse, en rappelant ici quelques principes fondamentaux qui avaient été largement oubliés et en soulignant là qu'une réforme nécessite des moyens, au moment même où on annonce la suppression de nombreux postes de fonctionnaires.

Le texte initial n'en restera pas moins comme une sorte de témoignage méritant de figurer au musée des textes anticonstitutionnels. Il est en effet remarquable d'avoir oublié autant de principes fondamentaux.

en cas d'échec d'une mesure alternative ou en matière de récidive légale. Le principe d'individualisation de la peine, que nous pensions être inscrit pour des siècles dans notre culture juridique, est écarté. juridique, est écarté. Les peines planchers, l'extension des amendes forfaitaires au-delà des contentieux de masse, le nouveau régime des réductions des peines sont autant d'illustrations du refus de la réalité pénale qui implique toujours un homme et des circonstances. Heureusement, notre rapporteur a redonné au juge un pouvoir d'appréciation grâce à une décision spéciale et motivée, c'est-à-dire grâce à une mesure qui sera l'exception, alors que la règle sera le refus de l'individualisation.

légalité. Vous avez en effet réussi cet exploit d'inventer une peine qui ne soit ni claire ni intelligible, en précisant qu'il fallait réprimer une manifestation d'adhésion ou de soutien à une organisation prônant la commission d'actes portant atteinte à des ressortissants français ou aux intérêts fondamentaux de la nation française.

serait évidemment incompatible avec l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel le port du bracelet électronique constitue bien une privation de liberté.

planchers, dont le bilan n'est pas fameux. En 2010, dans 62 % des cas éligibles, ces peines minimales ont été écartées par les juridictions répressives. En 2014, à la fin de la période, l'Union syndicale des magistrats

Cette proposition de loi a au moins pour mérite de montrer que, en matière pénale, les Républicains n'ont pas d'autre doctrine que le retour au passé et, finalement, le souci de plaire, sans se préoccuper des droits fondamentaux, sans évoquer les moyens qu'une telle proposition nécessite, sans s'inquiéter d'une justice forte et indépendante.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à quelques semaines de l'élection présidentielle, il est regrettable de débattre d'un texte portant sur des questions aussi importantes pour notre droit pénal. en effet peu probable que cette proposition de loi, signée par la majorité sénatoriale, soit examinée à l'Assemblée nationale d'ici à la fin

même que les conclusions de la mission pluripartisane pour « un véritable redressement de la justice », conduite par la commission des lois depuis juillet 2016, n'ont pas encore été rendues.

La volonté affichée de ce texte est- déjà, ai-je envie de dire -d'effacer ce qui a été fait, notamment en supprimant les mesures principales de la loi Taubira du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Ainsi, le coeur du texte repose sur le rétablissement des peines planchers et la suppression de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte, deux mesures pourtant destinées à encadrer davantage les condamnés et préparer leur réinsertion pour lutter contre la récidive. Par ailleurs, le quantum de peines aménageables est réduit, la compétence des juges de l'application des peines, limitée. Le texte développe également le recours aux procédures automatiques comme l'amende forfaitaire pour les délits correctionnels. Enfin, au-delà d'une volonté affichée de répression systématique, le texte traduit un mouvement de fond qui tend à évincer le juge du débat pénal ou, à défaut, à contraindre le contenu de ses décisions en battant en brèche le principe d'individualisation des peines, sans bien sûr aucune garantie corrélative d'indépendance des parquets. L'Union syndicale des magistrats a dénoncé devant la commission des lois les ressorts « démagogiques » d'un texte « à visée incarcératrice Étant donné l'importance des mesures envisagées, nous nous étonnons que cette proposition de loi n'ait pas été soumise pour avis au Conseil d'État avant son examen en commission, comme le prévoit l'article 39, alinéa 5, de la Constitution,

au président du Sénat de bien vouloir mettre en oeuvre cette disposition importante de notre Constitution à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, par courrier qui lui a été transmis hier. hier. Le travail du rapporteur François Pillet sur ce texte est révélateur des difficultés qu'il pose. Plusieurs propositions qui présentaient un caractère inconstitutionnel

Cependant, l'esprit du texte reste le même. Il s'agit, comme l'a dénoncé le Syndicat de la magistrature, « d'une nouvelle tentative pour introduire dans notre arsenal judiciaire des dispositions sécuritaires visant à incarcérer toujours plus En témoigne la volonté de créer de nouveaux « centres de rétention pénitentiaire » pour les détenus de brève durée. Cette vision du tout-répressif et l'aggravation des sanctions pénales pour la « petite délinquance » sont inadmissibles lorsqu'on lui oppose la « grande délinquance », financière par exemple, qui est pour sa part rarement sanctionnée par des peines de prison effectives en raison de multiples dispositions législatives ou réglementaires qui permettent d'y échapper. d'y échapper. Ainsi, certains et certaines parviennent à échapper à toute sanction et conservent un casier judiciaire tout à fait vierge, alors qu'ils encourent jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison. Et dans ce cas, mes chers collègues, on ne vous on ne vous entend guère vous émouvoir sur l'absence de fermeté et de sévérité de la justice. Pourtant, d'autres solutions que la création de nouveaux centres pénitentiaires existent pour lutter contre la surpopulation carcérale, comme faire de la détention provisoire une exception, et non la règle ! « C'est comme si la pire des situations devait peser sur des personnes n'ayant pas, ou pas encore, été condamnées », explique à ce sujet Jean-René Lecerf, qui préside la commission du Livre blanc sur l'immobilier pénitentiaire que vous avez installée la semaine dernière, monsieur le garde des sceaux. Ceux qui partagent les valeurs du progrès doivent avoir le courage de réaffirmer que la prison n'est pas la seule solution. Chacun ici dénonce le taux de récidive. Vous savez tous qu'il est de notre responsabilité de préciser les conditions de l'emprisonnement, y compris pour les délits mineurs. Notre attitude n'est pas laxiste, elle vise l'efficacité en dehors de l'émotion et de la démagogie. Donner la priorité aux peines alternatives, réorienter les peines vers la réinsertion, c'est une nécessité pour les victimes comme pour les coupables. En définitive, pour tendre vers une justice pénale efficace et humaine, il faudrait lancer un vaste chantier de réflexion et d'enquête sur les peines : leur sens, leur échelle et leurs modalités. Peut-être qu'il faudrait s'inspirer de ce qui a été fait en la matière depuis un certain nombre d'années dans les pays scandinaves, où le droit pénal est très avancé, comme en Norvège, où la criminalité est plutôt basse avec des taux de récidive très satisfaisants, à mettre en lien avec un traitement humain et individualisé des prisonniers. Mais il n'y a guère de mystère

Inutile de multiplier les textes, la justice pénale de notre pays ne sera efficace et humaine que lorsque ses moyens seront revalorisés et les magistrats augmentés. C'est pourtant tout le contraire que laissent présager les importantes suppressions de postes de fonctionnaires annoncées le candidat à l'élection présidentielle des Républicains. Sans surprise, et comme nous l'avons déjà dit en commission, nous ne voterons pas ce texte antinomique avec notre conception de la justice.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, il me semble opportun de considérer ce texte comme inopportun

égards à un texte d'opportunité électorale, ce dont personne ne doute dans cette assemblée. Soyons clairs : si vous gagnez l'élection, vous ferez pire ! Et si vous la perdez, nous ferons autre chose ... C'est d'autant plus dommage, monsieur le président de la commission des lois, que vous poursuivez une mission tout à fait intéressante et utile sur le redressement de la justice. Quelle cohérence peut-il y avoir

La seule explication, c'est que vous voulez essayer d'en tirer un profit médiatique à proximité de l'échéance électorale présidentielle. Je ne crois pas qu'il soit bon que les responsables politiques et les médias continuent d'intenter un procès injuste à la justice de notre pays, en particulier à la Cour de cassation.

des poussées médiatiques d'un certain nombre de médias nationaux. Les magistrats et les citoyens n'y comprennent plus rien et je crois qu'il faut davantage faire confiance aux magistrats. Certes, dans toute corporation,

Monsieur le président de la commission des lois, dans ce texte, il y avait manifestement plusieurs mesures peu conformes à la Constitution qui auraient justifié que vous appliquiez la jurisprudence que vous avez appliquée sur la Corse ! En conclusion, je crois que la justice mérite mieux. Elle mérite une loi de programmation préparée autour d'un large consensus politique, en concertation avec ceux qui la rendent, c'est-à-dire les magistrats.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes encore en début d'année et voilà déjà un nouveau texte qui réforme la justice. Et il ne manquera pas d'en venir d'autres après les élections J'ai recensé les textes consacrés à la justice depuis une douzaine d'années : nous en sommes à une vingtaine- j'en ai communiqué la liste précise au président de la commission des lois.

les magistrats n'ont pas les moyens d'exercer correctement leur mission. Notre justice est toujours insuffisamment dotée, eu égard à ses besoins

sans juge. Mais, parallèlement, d'autres réformes récentes accroissent les tâches des juridictions. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, les contestations des placements en centre de rétention administrative passent du juge administratif au juge judiciaire, en l'occurrence le juge des libertés et de la détention. Évidemment, si les questions budgétaires ne doivent pas nous interdire de réfléchir à des pistes d'amélioration, la question des moyens doit rester une préoccupation permanente, afin que telle ou telle mesure nouvelle ne vienne pas aggraver une situation qui, dans la plupart des juridictions, est déjà plus que préoccupante. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui est ambitieux, puisqu'il aborde presque tous les aspects de la politique pénale, depuis les mesures alternatives aux poursuites jusqu'à l'application des peines. Certaines de ses propositions sont la reprise de critiques anciennes formulées par notre commission. On peut citer la contrainte pénale, dont nous avions dit à l'époque qu'elle serait inutile et inefficace. Les faits nous ont donné raison, puisque, notre rapporteur l'a rappelé, les magistrats, parfaitement familiers du sursis avec mise à l'épreuve, ne se sont absolument pas approprié ce nouvel outil, quasi similaire, dont ils ne voient pas l'intérêt. Les statistiques parlent d'elles-mêmes depuis 2014, 2 000 mesures de contrainte pénale ont été ordonnées, contre 80 000 sursis avec mise à l'épreuve. Y renoncer aujourd'hui serait donc une mesure de bon sens. Je partage, avec notre rapporteur, le souci de renforcer l'effectivité de l'exécution des peines. Celle-ci est absolument essentielle pour la crédibilité de la réponse pénale. Comment justifier une exécution des peines plusieurs mois, voire un an après leur prononcé ? Nos concitoyens, confrontés à cette réalité, en sont ulcérés et ils ont raison. Cette proposition contient plusieurs dispositions qui concourent à améliorer l'exécution des peines ; nous les soutenons. La proposition de loi comprend également plusieurs mesures de simplification procédurale

Je tiens, enfin, à saluer le travail réalisé par notre collègue François Pillet sur ce texte. Comme d'habitude, il s'est montré précis, vigilant et constructif. Il a proposé, à juste titre, à notre commission de ne pas retenir plusieurs dispositions du texte initial qui lui paraissaient inopportunes, voire contre-productives. Suivant ses conseils, nous avons ainsi supprimé les articles 1 et 2, considérant notamment que l'automatisation de l'engagement des poursuites en cas d'échec d'une mesure alternative, contraire au principe au principe d'opportunité des poursuites, risquait d'avoir des effets contre-productifs et de réduire le taux de réponse pénale. Plus généralement, il a su éviter les et les caricatures. et les caricatures. Non, il ne faut pas laisser penser que certaines mesures de ce texte constitueraient une forme de défiance vis-à-vis des juges. Grâce aux modifications de notre rapporteur, que ce soit pour les peines planchers, la révocation du sursis ou la réduction des peines, le dernier mot reviendra toujours au juge.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi visant à renforcer l'efficacité de la justice pénale- sujet ô combien important, alors que la violence est omniprésente et au moment où le sentiment d'impunité gagne dans l'opinion publique Il faut dire que les différentes réformes mises en oeuvre par le Gouvernement- par exemple, la suppression de la contrainte pénale -ont contribué à alimenter le débat sur une justice à deux vitesses, avec la question des peines d'emprisonnement ferme de moins de deux ans qui, dans la plupart des cas, ne sont pas exécutées. C'est pourquoi, alors que se multiplient les actes délictueux

En effet, la justice est en crise et elle va mal. Les tribunaux sont engorgés, les procédures, longues, compliquées, reportées, et bon nombre de peines, non exécutées Pourtant, l'accès au droit est un pilier essentiel de toute démocratie et c'est la raison pour laquelle la justice doit être indépendante, efficace et accessible à tous. L'accumulation des lois désoriente les justiciables, l'instabilité de la législation complexifie la tâche des professionnels du droit et la surtransposition des directives européennes entraîne un surcoût financier. Si, en France, « nul n'est censé ignorer la loi », il faut bien reconnaître que peu la maîtrisent. Cette situation contribue à un sentiment d'insécurité de la part de nos concitoyens et alimente une forme de défiance

Ce domaine n'échappe pas à une nécessaire réforme et les axes retenus par ce texte vont dans le bon sens. En effet, renforcer l'efficacité des poursuites pénales, renforcer l'effectivité des alternatives aux poursuites renforcer le contenu de la réponse pénale constituent autant de mesures qui sont de nature à corriger l'image trop laxiste de l'appareil répressif et font apparaître la sanction plus clairement. Ainsi, les délinquants ne pourront plus échapper aux sanctions et les décisions auront valeur d'exemplarité. Je me félicite également du renforcement de la protection des mineurs et du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Là encore, ce sont des mesures qui complètent efficacement l'arsenal judiciaire et concourent à la sécurisation des populations, notamment des plus fragiles comme les mineurs. La nouvelle rédaction de la contrainte morale dans la qualification des infractions sexuelles était attendue depuis longtemps. Tout ce qui peut restaurer l'effectivité de l'exécution de la peine doit être mis en oeuvre par le législateur. Il est essentiel de redonner leur valeur d'exemplarité aux décisions de justice et du sens aux peines prononcées. Le nombre de peines de prison ferme non exécutées oscille actuellement entre 80 000 et 100 000. Par l'effet des réductions de peines automatiques et des mesures d'aménagement, la durée des peines exécutées est fortement réduite. Au 1 janvier 2017, 68 432 personnes étaient détenues en France. Parmi elles, combien de récidivistes ?

Actuellement, 19 498 personnes non encore jugées ou dont la peine est frappée d'appel sont incarcérées. La création de centres de rétention pénitentiaire à sécurité adaptée pour les détenus qui présentent une faible dangerosité et un risque d'évasion limité est un moyen efficace de lutter contre la surpopulation carcérale.

Même si la détention doit être dissuasive, elle doit être digne et humaine. Au-delà du sujet de l'immobilier pénitentiaire se pose le problème des procédures.

Cette proposition de loi va donc dans le bon sens. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail de notre collègue François Pillet, rapporteur de la commission des lois- commission présidée notre collègue Philippe Bas qui permet à ce texte de gagner en lisibilité et de tendre vers un objectif de confiance rétablie. Les articles qui la constituent répondent, d'une part, à l'exigence d'efficacité et, d'autre part, aux besoins des acteurs de la chaîne judiciaire pour agir plus sereinement. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons que nous réjouir des dispositions permettant de préciser l'intelligence avec une puissance étrangère et de compléter le délit d'entreprise individuelle terroriste. Cette réforme de la procédure pénale doit aider la justice à être plus simple, plus efficace, plus indépendante.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, la justice est malade et le malade est sous respiration artificielle ! Rarement autant d'experts et d'acteurs de la justice n'auront partagé ce constat. L'intérêt de l'initiative sénatoriale que nous examinons aujourd'hui est d'appréhender la question du bon fonctionnement de la justice dans sa globalité et du point de vue de son efficacité.

Chacun des six chapitres de la proposition de loi correspond à une étape de la procédure pénale : renforcer l'effectivité des alternatives aux poursuites ; renforcer l'efficacité des poursuites pénales et la capacité du procureur de la République à agir plus en amont dans la procédure renforcer le contenu de la réponse pénale ; restaurer l'efficacité de l'exécution de la peine prononcée ; renforcer la lutte contre le terrorisme ; renforcer la protection des mineurs. Concernant le chapitre IV visant à restaurer l'effectivité de l'exécution des peines, l'article 21 supprime la contrainte pénale, issue de la loi Taubira, et la libération sous contrainte, afin de restituer son efficience au sursis avec

phénomène à plusieurs facteurs, parmi lesquels l'augmentation du nombre de peines d'emprisonnement prononcées. Dans le même temps, il y a effectivement lieu de s'interroger sur l'efficacité du dispositif de contrainte pénale, mis en place en 2014 par Mme Taubira- et avec quelle assurance 2016, le bilan de cette mesure phare de la réforme pénale s'avère bien sombre. Il faut l'admettre, ce dispositif n'a jamais véritablement pris.

Quelles sont les raisons de l'échec de ce dispositif ? le sursis avec mise à l'épreuve, créé en 1958, qui a très largement les faveurs des juridictions répressives. Finalement, la contrainte pénale se distingue difficilement, par son contenu,

la question des moyens alloués à ces services est évidemment essentielle. En moyenne, un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation gère plus de cent dix dossiers

cette nouvelle usine à gaz mérite d'être supprimée, tout comme la libération sous contrainte. Tel est l'objet de l'article 21. Toute mesure dans ce domaine doit s'appuyer sur la sanction et la responsabilité individuelle. Elle doit combiner prévention, dissuasion, sanction et réinsertion, mais doit être fondée sur l'efficacité, la rapidité et la fermeté. Plus largement, le code de procédure pénale fait, aujourd'hui, de l'aménagement de la peine le principe et non l'exception.

Il s'agit donc de redonner toute sa place au sursis avec mise à l'épreuve, en renforçant l'efficacité du contrôle et de la prise en charge des personnes condamnées, sans pour autant grever davantage le budget. 22 de la proposition de loi prévoit la réintroduction des délégués bénévoles à la probation qui, pour les dossiers les moins lourds, viendront alléger la charge des agents des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

d'illusions ... La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

de mise en liberté rendue contrairement à ses réquisitions. Après avoir reçu notification d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions, le procureur de la République dispose de quatre heures pour, en même temps qu'il interjette appel, former un référé-détention, qui suspend temporairement les effets de l'ordonnance. La proposition de loi initiale prévoyait que ce référé-détention pourrait être introduit À introduit À la fin de l'information, la personne retenue- d'abord pendant quatre heures, puis pendant deux jours -l'aurait donc été sans que cette privation de liberté soit fondée sur un titre. Or le référé-détention est inapplicable en l'absence de titre initial de détention. C'est d'ailleurs ce que prend en compte la réécriture de l'article par la commission. Cependant, nous restons opposés à l'extension du référé-détention

pourrait s'appliquer aux ordonnances de mise en liberté « rendues par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, d'office, sur demande de mise en liberté, après renvoi devant le tribunal correctionnel ou après mise en accusation devant la cour d'assises ». Il pourrait du juge d'instruction disant n'y avoir pas lieu à saisine du juge des libertés et de la détention » et à celles « du juge des libertés et de la détention disant

Cette disposition, lourde de conséquences en termes de privation de liberté, participe à la volonté du « tout-carcéral » de la majorité sénatoriale. Le groupe écologiste s'y oppose fermement. Je rejoins donc nos collègues du groupe CRC, qui viennent de s'exprimer et qui demandent sa suppression. Quel

mercredi, un policier a été agressé à Corbeil-Essonnes, après qu'un autre de ses collègues l'eut été quelques jours auparavant par le jet d'un parpaing, avec une volonté criminelle clairement identifiée.

Il est intolérable et inacceptable que, dans notre pays, la couverture mobile soit aussi mauvaise, notamment dans les zones rurales.

La plateforme « France Mobile » est un sous-dispositif pour les territoires ruraux, que l'on finit par considérer comme sous-développés. C'est faux ! C'est inadmissible ! Il s'agit d'une vaste usine à gaz,

ce matin, conformément à la loi, vous présentiez le Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela a été l'occasion d'identifier les enjeux et d'établir une trajectoire budgétaire pour les années à venir. Nous nous félicitons des ambitions portées par ce rapport et, plus particulièrement, de la recherche d'une réelle mise en cohérence de plusieurs stratégies complémentaires. Nous saluons également la volonté de diplômer 60 % d'une classe d'âge, l'appui apporté à l'immobilier et à la politique de sites, ainsi que la revalorisation des traitements des enseignants-chercheurs et des personnels administratifs. Enfin, l'ambition de consacrer 2 % du PIB à l'enseignement supérieur et à la recherche, ainsi que 3 % à la recherche et développement, va réellement dans le bon sens. Dans le contexte actuel, cette question est malheureusement peu abordée dans les différents débats préélectoraux. L'exemple des dérives auxquelles on assiste aux États-Unis- gels de crédits, censure de chercheurs, mise au pas de la science de l'environnement et du climat -doit nous interpeller et nous conduire à placer ce sujet au coeur du débat politique, sans polémique inutile. Le Livre blanc retient qu'il faut faire de ce sujet un pilier majeur de notre développement socio-économique, pour lutter contre le chômage et la robotisation. Si nous en sommes convaincus, nous pensons que l'enseignement supérieur et la recherche doivent nous aider à appréhender la société de demain dans son ensemble. C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, le groupe écologiste vous interroge sur la place concédée à la transition énergétique, aux nouveaux modes de production agricole et à la santé dans la stratégie que propose le Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont nous espérons pouvoir débattre ici avant la fin de nos travaux. La

est un outil de pilotage stratégique sur cinq années du dispositif d'enseignement supérieur et de recherche. Toutefois, il est beaucoup plus qu'une obligation légale. Il est d'abord l'expression d'une conviction, que partagent nombre de

est ensuite l'expression d'une volonté, celle que notre pays demeure dans les toutes premières puissances mondiales en matière de diplomation, comme en matière de recherche, au moment où de grands pays annoncent des investissements massifs. La semaine dernière encore, les Britanniques décidaient de consacrer 4 milliards d'euros supplémentaires à la recherche pour les quatre années qui viennent ... Ce document est enfin une nécessité, alors que, d'outre-Atlantique, nous vient une contestation des bases mêmes de l'esprit scientifique,

Il mesure en outre, pour la première fois de manière indépendante, l'impact de l'investissement en matière de recherche et d'enseignement supérieur sur la croissance, c'est-à-dire un demi-point de PIB à l'horizon de dix ans. vous m'interrogez sur le développement durable, la transition écologique et d'autres thématiques. En 150 pages, il me semble que le développement durable est mentionné une cinquantaine de fois,

Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos cohortes aspirant à la liberté, envoyez-moi les rejetés de vos rivages, de ma lumière j'éclaire la porte d'or.

Presque 115 ans plus tard, les valeurs d'accueil et de solidarité américaines ne s'appliquent plus pour les ressortissants de sept pays du Moyen-Orient. Parce que M. Donald Trump, devenu locataire de la Maison-Blanche, a signé ce décret d'interdiction infâme, Irakiens, Iraniens, Yéménites, Libyens, Syriens, Soudanais et Somaliens ne sont plus les bienvenus sur le sol américain. Ce décret interdit pendant 90 jours toute entrée sur le territoire américain aux ressortissants de ces sept pays. Il bloque également, pendant la même période, les entrées de réfugiés en provenance de ces États. Face à cet acte, les réactions nationales et internationales ont rapidement couvert les quelques soutiens de la mesure, y compris de la part d'élus de la République française. La juge fédérale Ann Donnelly a partiellement annulé le décret. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a invité les réfugiés à opter pour le Canada, à défaut des États-Unis. Enfin, Mme Angela Merkel a donné une leçon de droit humanitaire à Donald Trump. La réponse de notre pays n'a pas été la plus rapide dans ce concert des réactions internationales, et beaucoup s'interrogent sur ce retard pris par la France. Nous pensons pour notre part, monsieur le Premier ministre, que la France a le devoir de faire entendre sa voix avec la plus grande clarté et la plus grande fermeté, au nom des valeurs humanistes qu'elle porte toujours dans le monde.

dans la maîtrise et la responsabilité, de renforcer les échanges de renseignements entre les grands services, ainsi que les coopérations en matière de lutte antiterroriste, et d'agir ensemble là où sont les foyers susceptibles de déstabiliser nos continents, comme nous le faisons au Levant dans la coalition. Pour que

Monsieur le ministre, l'action en faveur des jeunes était une priorité annoncée pour ce quinquennat, et de très nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement pendant ces cinq dernières années. Il fallait redonner espoir aux jeunes générations et leur préparer une meilleure place dans la société.

La majorité sénatoriale a tout fait pour empêcher l'adoption de ces mesures favorables à la jeunesse de notre pays, allant jusqu'à interdire le débat en votant une question préalable, puis à saisir le Conseil constitutionnel dès l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. avec cette loi, le Gouvernement renforce son action pour rassembler tous les Français autour des valeurs de la République. Cette loi contient des mesures innovantes pour la mixité sociale et pour la jeunesse. Elle crée les conditions de la généralisation d'une culture de l'engagement citoyen tout au long de la vie et renforce la priorité à la jeunesse portée par le Gouvernement depuis 2012. Je veux citer, en particulier, la création d'un congé d'engagement associatif pour les actifs bénévoles, la mise en place de la réserve civique tout au long de la vie, l'ouverture du service civique à de nouveaux viviers, pour atteindre l'objectif de 350 000 jeunes engagés par an à partir de 2018, la reconnaissance systématique de l'engagement dans les diplômes de l'enseignement supérieur, le financement du permis de conduire par le compte personnel de formation, le droit de publication et la majorité associative à 16 ans. Monsieur le ministre, toutes ces mesures sont importantes, concrètes et, surtout, très attendues par la jeunesse de notre pays. Aussi, pouvez-vous nous préciser le calendrier d'application de cette belle loi ? La

tout salarié du secteur public ou du secteur privé peut demander un congé de six jours pour se consacrer à son engagement bénévole associatif. C'est une manière de concevoir la démocratie dans notre pays. Autre progrès dont nous pouvons nous réjouir, il sera possible, désormais, de financer son permis de conduire grâce au compte personnel de formation. C'est là aussi un progrès très important, nombre de jeunes perdant des possibilités d'emploi parce qu'ils n'ont pas ce titre.

nettement inférieure à ses propres prévisions, lesquelles tablaient, chacun le sait, sur 1,4 % du PIB. D'après le ministre Sapin, ce chiffre aurait permis- il faut oser le dire

-économiques risquent de conduire directement au suicide de l'Union monétaire, tant vos résultats sont autant de manquements à nos engagements pour la convergence des économies de la zone euro

Reconnaissez, monsieur le sénateur, que, en un an, 110 000 chômeurs de moins sont inscrits à Pôle emploi. Vous pouvez dresser un bilan sur l'ensemble du mandat, ou sur le seul mois de décembre,

La situation, déjà délicate, s'aggrave progressivement : outre les 143 000 sans domicile fixe recensés par l'INSEE cette année, ce sont plus de 3 millions de personnes

Ce constat d'aujourd'hui est celui de plusieurs décennies d'inefficacité à fournir un logement décent à chacun. En moins de vingt ans, les prix de l'immobilier ont doublé et, depuis l'an 2000, les loyers des grandes agglomérations ont augmenté de 55 % en moyenne, deux fois plus vite que l'inflation. Aller plus loin dans l'encadrement des loyers, aller vers plus de transparence dans la construction et l'attribution de logements sociaux, aller vers plus d'hébergement d'urgence, voilà la démarche qui a été entreprise depuis cinq ans par les ministres successifs. J'ajouterai la diminution des nuitées d'hôtel, la lutte contre l'habitat indigne ou encore l'encadrement des loyers. À ce titre, je tiens tout particulièrement à saluer le travail et la dynamique entreprise par le Gouvernement en matière de logement, de lutte contre la précarité et l'exclusion dans l'habitat, de construction, d'urbanisme et d'aménagement foncier, ainsi que la politique en faveur du développement d'un habitat durable sur les territoires. Le Gouvernement a en effet veillé à la réduction des inégalités territoriales et sociales en matière de logement. Je pense notamment à l'instauration, par un décret ministériel de la ministre du logement, d'un sous-préfet dédié à la lutte contre l'habitat indigne, disposition mise en place par le biais de ma proposition de loi sur la lutte contre les marchands de sommeil et la lutte contre l'habitat indigne.

loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, promulguée le 27 janvier dernier, va améliorer la mixité sociale sur tous les territoires, tout en s'employant à améliorer le relogement des publics prioritaires. quelque 2 130 000 permis de construire qui ont été délivrés et 1 800 000 logements qui ont été mis en chantier. Quant aux logements sociaux, ils sont 130 226 à avoir été livrés en 2016, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2015.

Élisabeth Badinter déclarait il y a un an : « Il ne faut pas avoir peur de l'accusation d'islamophobie ». Elle proclamait ainsi son refus de céder au chantage antiraciste. Depuis lors, ce chantage n'a pas désarmé, bien au contraire ! Il y a quelques jours, c'est l'historien Georges Bensoussan qui était poursuivi pour provocation à la haine raciale. À l'origine de ce procès, un attelage d'un nouveau genre, le Collectif contre l'islamophobie en France et son cortège d'imprécateurs. Même la LICRA s'est solidarisée Animés d'une même fureur inquisitoriale, ils ont traîné en justice un historien de la Shoah qui serait coupable d'avoir dénoncé un antisémitisme devenu courant dans nombre de familles musulmanes. Le parquet l'a poursuivi. Peu auparavant, le philosophe et essayiste Pascal Bruckner a, lui aussi, comparu pour des reproches similaires. Dans son cas, la décision des juges a été une victoire de la liberté d'expression contre l'intimidation islamiste. Il y a quelque chose de réconfortant à constater que la justice n'est pas dupe de la stratégie de certains groupes identitaires ! Si cette décision est le fruit de la sagesse, on peut, en revanche, s'étonner de la frilosité du Gouvernement, que l'on a si peu entendu sur ce sujet. également s'étonner de la situation de certains « territoires perdus de la République », où l'enseignement de la Shoah est devenu impossible et où l'idéologie de l'opprimé et du relativisme installe l'idée que les coupables de tous les maux sont la République et la France. Monsieur le garde des sceaux, ne croyez-vous pas qu'il est temps de condamner fermement le discours selon lequel la France serait islamophobe ? Ne croyez-vous pas qu'il est temps de soutenir nos enseignants dans leur lutte pour la liberté d'expression et le droit d'enseigner l'histoire et les sciences naturelles et, finalement, de défendre, là aussi, la République ? N'est-il pas temps pour le Gouvernement de le dénoncer, pour défendre la République contre ses fossoyeurs ?

ont reçu une circulaire de politique pénale que j'ai signée en juin 2016, dans laquelle je réaffirme comme priorité la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Je puis comprendre la volonté polémique, mais je ne la crois assise sur aucun fait

mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, Mayotte connaît depuis le mois de novembre dernier la période de sécheresse la plus alarmante de son histoire en raison d'un fort déficit pluviométrique et d'une saison des pluies retardée. Les deux retenues collinaires alimentant l'ensemble de l'île en eau potable sont presque vides. Dans le sud, la retenue contient, aujourd'hui, un peu plus de 15 % de sa capacité et à peine plus de 20 % dans le nord. Des mesures de restrictions ont été prises pour limiter la consommation et, depuis la fin du mois de décembre dernier, un dispositif de coupures d'eau deux jours sur trois a été mis en place dans huit communes du département. La rentrée scolaire a même été reportée du 9 au 12 janvier dans la grande majorité des établissements scolaires des communes concernées par ces coupures, le temps de préparer des approvisionnements. De manière générale, à Mayotte, l'eau douce est une denrée rare, difficile à gérer entre pression migratoire excessive, insularité et augmentation de la consommation en eau des ménages. Aussi, je souhaiterais savoir quelles mesures d'urgence le Gouvernement entend prendre, en concertation avec le syndicat des eaux et les collectivités de Mayotte, pour remédier à cette pénurie dramatique, dont il est inutile de préciser les conséquences en matière de risque sanitaire. Par ailleurs, pour prévenir ce type de situation, ne pourrait-on envisager de mettre en oeuvre une grande politique de sensibilisation à la protection de l'environnement à l'attention de la population mahoraise ? Il est également impératif qu'une troisième retenue collinaire, en projet depuis plus d'une décennie, soit effectivement construite pour tenir compte des réels besoins en eau des Mahorais. La

avec lesquels la ministre des outre-mer est en contact quotidien, réalisent actuellement un suivi de l'évolution de la situation, en lien avec le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte et avec l'association des maires. rampes d'eau garantissant l'accès à l'eau potable ont été installées et plusieurs mesures prises par l'État depuis la fin du mois de novembre dernier ont permis de prolonger l'accès aux ressources existantes jusqu'à la fin du mois de mars.

qui permettront d'injecter cette eau dans le réseau de Mayotte. Il faudrait également raccorder le réseau du nord de l'île avec le réseau du sud. Le ministère des outre-mer est aussi particulièrement attentif à la situation des écoles, des collèges et des lycées. Nous travaillons pour que soit garanti l'accès à l'eau des élèves et des enseignants. Au-delà de l'urgence, il faut voir que, à moyen et à long terme, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Un travail de pédagogie va être mené pour diffuser une véritable culture de l'économie d'eau

La séance est reprise. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 8 février 2017, après l'examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain,

sur le projet de loi ratifiant les ordonnances du 14 mars 2016, relative à la partie législative du code de la consommation, et du 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs, initialement inscrites le jeudi 9 février. Le Gouvernement a également demandé l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 15 février 2017 des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à l'autoconsommation d'électricité et relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, ou de sa nouvelle lecture, après l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, ou de sa nouvelle lecture. Acte est donné de ces demandes. La commission des lois se réunira pour examiner le rapport sur la proposition de loi visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété le mercredi 1 février matin.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et en application de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, M. le Premier ministre, par lettre en date du 30 janvier 2017, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission du Sénat compétente en matière d'énergie sur le projet de nomination de M. Jean-François Carenco aux fonctions aux fonctions de président du collège de la commission de régulation de l'énergie. Cette demande d'avis a été transmise à la commission des affaires économiques. Acte est donné de cette communication. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et en application de l'article L. 2312-2 du code de la défense, M. le Premier ministre, par lettre en date du 31 janvier 2017, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission du Sénat compétente en matière de défense sur le projet de nomination de M. Jean-Pierre Bayle aux fonctions de président de la commission du secret de la défense nationale.

L'article 6 élargit le domaine de l'amende forfaitaire aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l'exception des infractions contre les personnes, qui sont couvertes par le livre II du code pénal. Cette disposition est contraire au principe d'individualisation des sanctions en matière délictuelle. Elle consacre en effet une nouvelle procédure automatique et rapide, qui ne permet pas l'expression des droits de la défense. Cela porte atteinte au principe du débat contradictoire et à celui de la séparation de la poursuite et du jugement. En outre, comme en témoigne l'extension de l'amende forfaitaire à certains délits routiers, adoptée dans la loi de modernisation de la justice du XXI siècle, cette disposition affaiblit la force de la sanction pénale.

irrégulier. Depuis lors, les conseils juridiques, ainsi que les prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux ne peuvent plus être poursuivis lorsqu'il s'agit d'une action humanitaire envers des personnes en situation irrégulière.

? Cet amendement vise à étendre le champ de l'immunité pénale en matière d'aide au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire français. L'aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France est constitutive d'un délit, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. toutefois pas incriminables les actions d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, soit lorsqu'elles sont le fait d'un proche de la personne étrangère, soit lorsqu'elles sont effectuées dans un but humanitaire. À mon sens, les situations mentionnées dans l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Certes, le transport n'est pas spécifiquement mentionné, mais, dans l'absolu, rien ne paraît empêcher qu'il entre dans ces catégories dès lors qu'il vise à préserver la dignité ou l'intégrité de

par l'article 131-21 du code pénal, qui porte sur la confiscation des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

concernant les personnes morales que sont, notamment, les sociétés civiles immobilières, méthode utilisée par les marchands de sommeil les plus attentifs aux décisions de justice. Cette confiscation n'est malheureusement que trop peu utilisée par les magistrats du siège ou du ministère public, alors qu'elle constitue, en complément des sanctions financières,

quelques dizaines de minutes. Une telle disposition est destinée à éviter qu'un détenu comparaissant libre ne prenne la fuite entre la fin des plaidoiries et le prononcé de la peine, ce qui participerait à la décrédibilisation de l'action de la justice.

De plus, la réintroduction des peines planchers porte atteinte au principe constitutionnel d'individualisation des peines et affaiblit le pouvoir d'appréciation du juge.

en cas de récidive : nous irions plus loin encore que le législateur de 2007 ! Il faut rappeler que les études actuellement disponibles sur les effets des mesures de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive ne permettent pas de conclure qu'elles auraient eu un effet déterminant sur la baisse de la récidive ou de la délinquance.

prononcées en cas de récidive, qui demeure autour de 94 %, comme le révélait l'étude d'impact de la loi de 2014. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article, qui, en rétablissant un dispositif n'ayant pas fait ses preuves, introduit une énième et inefficiente

caractère plus humain, qui tient compte de la personnalité et de la situation du condamné. De plus, l'affaiblissement de l'aménagement des peines s'oppose aux recommandations du Conseil de l'Europe et des règles pénitentiaires européennes, qui considèrent que la peine privative de liberté ne doit être que

l'amendement n° 10. Cet article avait pour objet initial de rétablir la révocation automatique et intégrale du sursis simple, supprimée par la loi Taubira du 15 août 2014. Même si les modifications apportées en commission par M. le rapporteur vont dans le bon sens, en permettant au juge de faire obstacle par une décision spéciale et motivée à la révocation automatique du sursis, les dispositions prévues continuent à nuire à l'individualisation des peines, principe à valeur constitutionnelle.

le mécanisme proposé nuit toujours à une appréciation fine et individualisée de la situation de la personne condamnée, ainsi que, par conséquent à l'efficacité de la sanction pénale. Par ailleurs, le texte ne rétablit pas la possibilité qui était auparavant ouverte à la personne condamnée de demander, lorsque la juridiction du jugement n'avait pas expressément statué sur une dispense de révocation du sursis, de bénéficier ultérieurement de cette demande. Le Gouvernement émet donc

très fréquemment adoptée par les juridictions, lesquelles refusent souvent la confusion des peines lorsque les infractions sont de nature différente. De plus, et c'est un leitmotiv cette après-midi, il est essentiel de souligner que, là encore, nous avons veillé à préserver le pouvoir d'appréciation des juges, qui auront la possibilité

d'office par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de sa dernière. Selon nous, cet article limitera de nouveau le pouvoir d'appréciation des juges et rendra encore plus automatiques les différentes peines, ce à quoi nous sommes opposés.

Néanmoins, contraindre les magistrats à relever d'office la récidive au stade de la poursuite et du jugement, sous réserve de l'opportunité des poursuites par le parquet, et à émettre une décision spéciale et motivée pour la juridiction

Le Gouvernement considère que la nouvelle répartition des compétences est de nature à alourdir très fortement la charge de travail des juridictions de l'application des peines et risque par conséquent de retarder les aménagements de peine et de nuire à la prise en charge des longues peines. En outre, cela ne paraît pas utile au regard de la possibilité que le juge d'application des peines a de renvoyer le dossier vers le tribunal de l'application des peines s'il l'estime nécessaire, renvoi qui s'opère en pratique au regard de la complexité du dossier

prévu devienne le seul régime de réduction de la peine. Il faut rappeler que le régime des crédits de réduction de peine a été instauré par la loi pénitentiaire

Par ailleurs, la question de l'accroissement du budget reste en suspens si ces suppressions sont mises en oeuvre. Les dépenses devraient plutôt être réorientées pour rendre efficaces ces aménagements de peine, car, à la différence de l'ancien sursis mise à l'épreuve, la contrainte pénale exige un suivi intense des condamnés et des renforts supplémentaires en conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, une justice efficace et humaine est à ce prix, et c'est une nécessité pour notre société.

disposition phare de la loi Taubira. Nous l'avons défendue, considérant que cette mesure, qui se déroule en milieu ouvert, est une peine à part entière, une peine dont la finalité est de responsabiliser et de réinsérer le condamné dans notre société. Nous souhaitions d'ailleurs avec force que cette nouvelle peine trouve rapidement toute sa place dans le système pénal, qu'elle soit véritablement appliquée et ne soit pas considérée par les magistrats comme une simple mesure de substitution au sursis avec mise à l'épreuve. Sa mise en application n'est probablement pas totalement satisfaisante à ce jour, mais nous continuons d'être favorables à cette mesure et nous nous opposons tout naturellement à sa suppression. La parole

de notre discussion. La contrainte pénale résume à elle seule toute la politique pénale de ce quinquennat. Nous avons tout d'abord des objections de principe très fortes à l'égard de cette politique, dont, avec la contrainte pénale, le principe devient l'alternative à la prison, et l'exception, la prison. À l'inverse, nous voulons une politique où le principe est la prison, et l'exception, l'alternative à la prison. Cette démarche, qui n'est pas que symbolique,

d'affirmer nettement l'exigence de la punition et de la sanction. Le deuxième élément pour lequel il faut renoncer à cette contrainte pénale, et non simplement la laisser dépérir d'elle-même alors que les juges ne la prononcent pas, est son échec

par an en moyenne face à 108 000 peines de prison -, permettent de mesurer l'inanité de ce dispositif, qui est massivement rejeté par les magistrats.

La contrainte pénale est une mesure beaucoup plus répressive. Que l'on cesse donc, monsieur le président de la commission des lois, de laisser accroire qu'il y aurait une droite répressive et une gauche laxiste. Ce n'est pas vrai

Comme l'exprime le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, M. Jean-Marie Delarue, « l'efficacité de la prison réside moins dans le jour de l'entrée que dans le jour de sortie du condamné ». S'il est des économies à ne pas faire lorsque l'on cherche à lutter contre la récidive, c'est donc dans l'accompagnement des probationnaires. Depuis une trentaine d'année, cette mission d'accompagnement s'est considérablement professionnalisée, en bonne intelligence avec le milieu associatif, qui assure une fonction support importante. nous craignons que la réintroduction de bénévoles ne casse cette dynamique de professionnalisation, qui est, vous l'avez compris, essentielle. Pour cette raison, nous proposons la suppression de l'article 22 de la proposition de loi. Quel est l'avis de la commission ? Loin de moi

ne nuit pas à l'apport du monde associatif et bénévole et lui permet, dans des conditions déterminées, d'apporter un soutien ponctuel aux équipes sur des missions limitativement énumérées.

23 veut restaurer l'effectivité de l'exécution de la peine et lutter contre la surpopulation pénitentiaire en définissant un nouveau type d'établissement pénitentiaire pour les détenus condamnés à des peines courtes et « considérés comme peu dangereux, ne risquant pas de s'évader et dont la peine restant à subir serait inférieure à un an

alors que les conditions de vie dans les maisons d'arrêt, dont le taux d'occupation est de 137 %, ne cessent de se dégrader. Et nous ne parlons pas de la hausse continue du nombre de détenus encore non jugés- presque 19 500 prévenus janvier dernier. Cette proposition de loi qui promet de rendre la justice plus répressive ne fera donc qu'accentuer le problème. Je le répète avec force : lutter contre la surpopulation carcérale ne consiste pas à créer de nouveaux centres de rétention, comme le suggère cet article. Un moyen simple de désengorger les prisons existe. Il consiste à faire de la détention provisoire une exception et non la règle, comme je l'ai déjà souligné lors de la discussion générale.

doter d'établissements dont le niveau de sécurité est largement allégé, puisqu'il correspond à des peines et à des personnalités qui, ne présentant pas de dangerosité particulière, ne nécessitent pas un arsenal

une nouvelle dérogation, un nouvel amoindrissement de cette réparation générale. M. le rapporteur propose notamment d'exclure la réparation dans les cas où « l'information judiciaire au cours de laquelle a été ordonnée la détention provisoire a fait l'objet d'une annulation et qu'une nouvelle enquête ou une nouvelle information judiciaire a été ouverte sur les mêmes faits.

les détentions provisoires ordonnées dans le cadre de procédures annulées, mais pour lesquelles une nouvelle enquête ou une nouvelle information judiciaire a été ouverte pour les mêmes faits. Imaginons que, à la suite de cette nouvelle enquête ou de cette nouvelle information judiciaire,

Le Gouvernement a bien noté le changement apporté par la commission des lois, qui n'a pas suivi le texte initial et qui a prévu d'exclure la réparation en cas d'annulation suivie d'une nouvelle enquête ou instruction.

! Deuxièmement, je veux redire, eu égard aux propos qui ont été tenus précédemment par un certain nombre de collègues d'autres groupes, qu'il ne s'agissait pas ici d'évoquer de quelque manière que ce soit de nouvelles infractions, de nouveaux quanta de peines ou l'augmentation de quanta de peines encourues pour des infractions commises.

laissant toujours, et de façon permanente, au juge la capacité de pouvoir décider autrement. Il est évident que l'individualisation de la peine reste le principe principe fondamental. Demain, n'importe quel magistrat pourra décider de ne pas appliquer un sursis, de modifier un sursis avec mise à l'épreuve, voire de ne pas appliquer une peine plancher en cas de récidive pour une peine encourue de plus de cinq ans. C'est essentiel. ans. C'est essentiel. Par ailleurs, nous sommes favorables au fait que nous puissions trouver des solutions en matière carcérale. Nous l'avons déjà dit de façon très claire, avec les éléments que nous avons donnés.

les gouvernements que nous soutenons ont créé de nombreux postes, alors que les gouvernements précédents en avaient supprimé. Nous voulons donner les moyens à la justice, et nous le faisons. Mais le débat principal

soutenons et que nous avons soutenues au cours de ces cinq années, pour une justice qui soit à la fois ferme, exigeante et humaine. Monsieur le président, mes chers collègues, la priorité à la réinsertion, la mise en place de peines alternatives à l'incarcération, l'abrogation des peines plancher, toutes ces mesures que nous avons défendues sur ces travées dans un récent passé ont vocation aujourd'hui à être supprimées, tout au moins par le Sénat. De surcroît, il est certain que les dispositions de la présente proposition de loi auront un impact tant sur la charge et l'organisation des juridictions de notre pays que sur les établissements pénitentiaires. La plupart d'entre eux étant déjà exsangues, il est impensable d'adopter un tel texte sans garantie aucune concernant le budget alloué à la justice. Les déclarations du candidat de la droite à l'élection présidentielle, soutenu par nombre des auteurs de ce texte, envisageant la suppression de 500 000 emplois publics, sont alors loin d'être rassurantes. rassurantes. Parce que nous considérons qu'il s'agit là d'un texte d'affichage à destination des électeurs de droite, le groupe écologiste votera

J'assume pleinement, en revanche, cette réalité que le Sénat est une assemblée permanente de la République

dans l'hypothèse de l'alternance, d'avoir un texte prêt pour que la nouvelle Assemblée nationale, au mois de juin prochain, puisse l'adopter immédiatement.

mais il va émettre un signal nécessaire, celui de la sévérité de la lutte contre la délinquance. Monsieur Sueur, nous avons un bilan des peines planchers. Les magistrats se sont sentis libres se sont sentis libres : dans plus de la moitié des cas, ils n'ont pas prononcée la peine plancher. C'est dire ! En revanche, le quantum des peines, tout le temps que la peine plancher a été applicable, a été augmenté en moyenne de six mois. Cela signifie que les magistrats nous comprennent très bien, mes chers collègues : nous leur demandons une plus grande sévérité, mais nous ne leur demandons pas de renoncer à leur office. Jamais !